Je veux ici de nouveau saluer les sapeurs-pompiers pour leur bravoure et pour leur dévouement. Je veux saluer nos agriculteurs et les nombreux citoyens qui ont aidé lors des feux dévastateurs de cet été. Ce que nous a appris 2022, c'est que désormais plus aucun territoire n'est épargné par le réchauffement climatique et que les incendies peuvent frapper même au nord de la Loire.

Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne. Nos moyens doivent être suffisants face à cette situation, qui s'annonce récurrente. Un certain nombre de mesures ont été mises en place depuis le mois d'octobre dernier.

et plus de la moitié sont liés à des imprudences- une étincelle, un mégot, un barbecue. Au-delà de la prévention et de la météo,

réplique. Merci, monsieur le ministre, pour vos précisions et vos réponses. Vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur notre territoire est une préoccupation principale de nos maires, qui sont en première ligne. Ils ont besoin de notre soutien. Les annonces que vous faites, notamment sur la prévention, sur le rapprochement des moyens aériens, sur le fonds vert, sur les sentiers, sont une excellente nouvelle. Vous pouvez compter sur le Sénat pour être à vos côtés et améliorer encore les dispositifs annoncés

fin de vie pour le pavillon individuel ; fin de vie pour les investisseurs dans l'immobilier ; fin de vie pour les emprunteurs modestes. Vous avez réussi l'exploit d'annoncer un plan de relance

rien sur les terrains, rien pour l'investissement et rien pour solvabiliser. Alors, madame la Première ministre, à quand le second plan, le vrai plan de reconstruction pour la France ?

je m'inscris profondément en faux contre tout ce que vous avez affirmé, et je m'étonne que vous soyez à ce point conservateur. D'abord, le CNR a été un succès. Il a permis de mobiliser plusieurs centaines d'acteurs du logement, dans des proportions

employant de nouvelles méthodes pour que les services des domaines et les services fiscaux puissent mieux évaluer le prix des terrains. Je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Conseil national de la refondation du logement était celui de tous les espoirs. Bénéficiant Bénéficiant d'une concertation inédite, d'un engagement total de la part de l'ensemble des acteurs du logement et fort de plusieurs centaines de propositions, le CNR devait constituer un tournant ambitieux pour notre politique du logement face à une crise sans précédent. Pourtant, il a tout d'un rendez-vous manqué. Les acteurs du logement sont unanimes : le compte n'y est pas. Pis, l'heure est à la désillusion et votre déni ne change pas le résultat. La politique du logement ne semble manifestement destinée qu'à être une variable d'ajustement budgétaire. Si l'on fait le bilan comptable de ce CNR, c'est plus de 2 milliards d'euros en moins pour la politique du logement. Ce n'est pas acceptable : c'est la refondation du logement que l'on attend ! « Le CNR n'était pas une fin en soi », a déclaré Olivier Klein. Pouvez-vous nous assurer qu'il est au moins le début de quelque chose ? Pouvez-vous nous dire si, dès le début du mois de juillet, des annonces seront faites pour le logement et si un plan d'ampleur sera enfin annoncé pour répondre à la colère non apaisée du monde

La Première ministre a donné rendez-vous, à la fin du mois de juin, à l'ensemble des ministres concernés et à la Caisse des dépôts et consignations pour aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Au cours de ces dernières semaines, et ce sera officialisé dans les prochains jours, nous avons établi une nouvelle convention quinquennale avec Action Logement, votée à l'unanimité par les partenaires sociaux.

avec l'ensemble des partenaires sociaux ? Vous savez également que la remise à plat d'une partie de la fiscalité sur la location, souhaitée par certains, a vocation à être examinée avant le début de la période budgétaire- il s'agit, là aussi, d'une annonce de la Première ministre. Je vous demande de prendre ce point d'étape pour ce qu'il est

les propositions issues du CNR laissent de trop nombreuses questions en suspens et nous avons besoin de réponses fortes. En dehors des métropoles, point de salut réponse apportez-vous aux besoins des territoires qui ne sont pas en zones tendues ? Comment accéder à la propriété en dehors des métropoles ? Quel parcours résidentiel pour les 2,4 millions de demandeurs de logement social ?

PTZ recentré, Pinel supprimé ... Pouvez-vous nous assurer que l'accession à la propriété restera une opportunité offerte au plus grand nombre et non un privilège accordé à quelques-uns ? du statut du bailleur privé ? Où et quand

4,1 millions de mal-logés ; 2,4 millions de ménages en attente d'un logement social. Le Val-de-Marne vient de franchir le cap des 100 000 demandeurs de logements. Dans le même temps, 5,7 millions de personnes consacrent plus de 35 % de leur revenu au logement ... Deux mots me viennent : souffrance et irresponsabilité.

si le logement coûte 38 milliards d'euros par an au budget de la Nation, il rapporte 88 milliards ! Dès lors, comment expliquez-vous que la part du PIB consacrée au logement n'ait jamais été aussi faible qu'en 2021 avec 1,5 % ? Un record jamais atteint

plus de 6 millions d'euros dépensés chaque soir. Oui, il faut continuer d'accompagner le logement social. Ce n'est pas un bâton de maréchal, mais je suis fier d'être un fils du logement social et d'en avoir occupé un longtemps au début de ma carrière d'enseignant. ! Il faut soutenir le logement social. C'est ce que nous avons fait en plafonnant l'augmentation du taux du livret A. Il faut soutenir le logement social dans sa capacité à rénover. Là encore, nous avons fait une annonce importante sur la seconde vie dans le cadre de rénovations lourdes, ce qui permettra

: gel immédiat des loyers, avec une compensation pour les bailleurs sociaux ; généralisation de la TVA à 5,5 % pour la construction de tous les logements sociaux ; généralisation des aides à l'accession sociale à la propriété, mais également interdiction de toutes les expulsions sans solution de relogement ; revalorisation immédiate des APL en tenant compte de l'inflation et de l'indice de référence des loyers ; plafonnement des prix de vente des logements en zone tendue ; plus grande taxation des plus-values immobilières pour financer le Fonds national d'aide au logement et inciter à baisser les prix de vente

ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, la grève des personnels de l'enseignement primaire dure depuis cinq semaines, voire six, à Wallis-et-Futuna, dans l'indifférence presque totale. Les grévistes sont déterminés à continuer le mouvement, parce que l'État les traite différemment. Voilà cinquante-quatre ans qu'ils assurent une mission de service public sans reconnaissance de l'État. Pourtant, une ordonnance du 15 février 2006 étendait à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française l'application de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Wallis-et-Futuna a été délibérément exclu

nos maîtres sont titulaires d'une licence des métiers de l'enseignement. Ils sont agréés par l'État et signent un contrat de travail avec le vice-rectorat, qui les gère et les paie directement. Monsieur le ministre, vous en conviendrez, la demande des grévistes que leur soit reconnu le statut d'agent public de l'État dès la rentrée 2024, avec tous les avantages liés, est parfaitement légitime. Les enseignants, à Wallis-et-Futuna, sont des citoyens français. Nos enfants sont des enfants de la République et doivent retourner en classe.

vous m'interpellez au sujet des maîtres et maîtresses de Wallis-et-Futuna, qui sont en grève depuis le 2 mai pour des raisons salariales. Je rappelle qu'à Wallis-et-Futuna les enseignants du premier degré sont des agents de droit privé, l'enseignement est concédé à l'enseignement catholique. Ces professeurs sont donc employés par la direction de l'enseignement catholique. Néanmoins, l'État assure leur rémunération, à hauteur de 4 500 euros brut mensuels, sans compter les primes. En outre, ces enseignants sont recrutés à bac+2, contrairement à la situation ordinaire

proposé des augmentations de rémunération. J'ai également donné mon accord pour que des groupes de travail se mettent en place afin de comparer la situation des maîtres et maîtresses de Wallis-et-Futuna avec leurs collègues de Nouvelle-Calédonie et d'étudier la possibilité de leur permettre d'accéder au statut d'agent public de l'État. Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous suivons de près la situation des quelque 150 maîtres et maîtresses concernés

Monsieur le ministre, le logement va mal. C'est un secteur en crise. Tous les indicateurs sont à la baisse : ventes de logements, mises en chantier, nouveaux permis de construire. Dans le même temps, on compte plus de 2 millions de personnes en attente d'un logement social : un record Après plus de six mois de travail, d'échanges et de concertations, les attentes étaient fortes. Mais lundi soir, lors de la conclusion du CNR Logement, la montagne a accouché d'une souris. La colère du secteur est à la mesure de sa déception face à un plan jugé minimaliste et imprécis, qui n'a conservé que très peu de ses propositions. Les deux copilotes du CNR Logement, les acteurs de l'immobilier, de la construction et de la solidarité, tous se sentent méprisés par le Gouvernement. Monsieur le ministre, il faut une impulsion forte pour répondre à la crise du logement. Pourquoi n'avez-vous toujours pas pris la mesure de ses conséquences économiques et sociales ?

Artigalas, comme cela a été rappelé plusieurs fois, y compris par vous-même, le CNR a été un moment extrêmement important de mobilisation et de travail des acteurs du logement. Il est tout sauf un point final : c'est un moyen de réfléchir à de nouvelles méthodes de travail sur lesquelles nous allons nous appuyer pour la suite.

nous avons décidé de multiplier par deux l'accès à Visale, notamment dans le cadre des accords que nous avons avec Action Logement. Là encore, Visale est une mesure de protection du pouvoir d'achat : c'est la caution de ceux qui n'ont pas de caution. Passer de 1 à 2 millions de Visale est donc extrêmement important et extrêmement utile pour nos concitoyens. Notre priorité est

en matière de foncier ? Rien n'a été fait pour rendre un peu d'autonomie fiscale aux élus ni pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété dans les territoires qui les ont vus naître. Aucune mesure n'a été prise non plus pour relancer la dynamique de la construction, perdue depuis 2017. Où est la refondation promise ? Le ministre délégué chargé des comptes publics a déjà annoncé que le secteur du logement subirait subirait une nouvelle baisse dans le budget 2024. La crise du logement s'aggravera, et ce sera à cause de votre inaction

Dans cette période émaillée de nombreuses crises, l'augmentation des tensions et le recours à la violence sont des signaux d'alerte à considérer avec une immense gravité.

J'y mesure également la méconnaissance de nos institutions et de notre fonctionnement démocratique. Tout cela va de pair avec une moindre compréhension de la décision politique et, de ce fait, avec une moindre acceptation des lois et des institutions. Ce défi démocratique, nous devons le relever. Au-delà des dispositifs déjà mis en place, qui relèvent de mesures davantage curatives que préventives, le groupe RDSE, avec notre collègue Henri Cabanel, a engagé un travail collectif pour développer le sens de l'engagement et la culture citoyenne. Ses propositions visent à permettre à chacun de trouver son rôle et sa place dans une société apaisée et de s'inscrire dans un projet commun, avec des références partagées. Au sein de ces propositions, l'éducation est une priorité, car l'ignorance est le terreau de la défiance et l'école le lieu où sont formés les futurs citoyens. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour mettre en place une véritable culture citoyenne à l'école ? La parole

celle de l'avenir de notre République et de notre démocratie. L'enseignement moral et civique, auquel vous faites allusion, fait partie des enseignements obligatoires dispensés du

Écoutons Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, qui confirment l'absolue nécessité de réorienter les financements publics vers tout ce qui rend notre société plus durable et résiliente. Écoutons les experts et les élus, dont les écologistes. Ils vous interpellent pour que les collectivités soient soutenues. Plus de 25 milliards d'euros par an doivent être mobilisés à leur niveau pour amortir les chocs annoncés liés à l'augmentation des températures de 4°C en France. Monsieur le ministre, nous n'avons plus le choix. Il faut faire en dix ans ce qui ne l'a pas été en trente. C'est un changement d'échelle et d'enjeu. Tous les leviers doivent être activés sans attendre et sans fléchir. les plus riches doivent-ils être mis à contribution, d'abord parce que ce sont les plus pollueurs, ensuite parce que les 378 ménages les plus aisés sont ceux qui payent le moins en proportion de leurs revenus, d'après la note de l'Institut des politiques publiques publiée hier, enfin, tout simplement, parce que la transition écologique doit se faire dans la justice sociale. Monsieur le ministre, comment allez-vous financer la transition et l'adaptation de notre pays au bouleversement climatique ? ? Vous dites non à un impôt vert exceptionnel sur le patrimoine financier des 10 % les plus riches. Vous dites non également à un endettement pourtant légitime afin de faire face à la gravité exceptionnelle de cette crise climatique. Monsieur le ministre, à quoi dites-vous oui ?

Si l'écologie devient le prétexte pour interdire et pour taxer, nous renforcerons l'impopularité de ces mesures auprès d'une partie de la population et nous nous éloignerons de nos objectifs. L'enjeu, monsieur le sénateur, est non pas la transition d'un impôt, mais la transition fiscale.

Monsieur le ministre, je vous remercie de me répondre par des questions ... Pour la crise de la covid-19, vous avez mobilisé sans compter, et c'était heureux ! Pour la crise climatique, c'est non, et cela nous choque. Monsieur le ministre, si la dette financière est un sujet sérieux et la transition fiscale une nécessité, commencez par l'ISF climatique, qui est

relèvent de la fonction publique hospitalière et ceux qui exercent dans des établissements privés ou privés à but non lucratif. En effet, en juillet 2022, vous avez décidé une majoration exceptionnelle de certaines indemnités horaires, notamment celles du travail de nuit et des heures supplémentaires, majoration qui est reconduite jusqu'au 31 août 2023. Ces majorations sont accordées aux professionnels des hôpitaux publics. Elles représentaient 531 millions d'euros en 2023 et 760 millions d'euros cumulés en 2022, versés aux 929 000 personnes du secteur public hospitalier, hors personnel médical. Ces majorations ne concernent que la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des professionnels des établissements privés et associatifs, qui sont au nombre de 284 000, alors qu'ils remplissent les mêmes missions et répondent des mêmes modalités de financement et de régulation de leurs activités. La situation de notre système de santé appelle à la mobilisation de tous, pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. La crise sanitaire a montré que des synergies étaient possibles entre les établissements de santé de différents statuts. Cet esprit de la covid-19 doit être préservé. Il passe par la reconnaissance de l'ensemble des professionnels de santé de tous statuts, soumis à de fortes tensions dans un contexte de pénurie des ressources humaines. alors que nous avons besoin de la mobilisation de tous, comment expliquer ce traitement inéquitable et comment comptez-vous être la garante de l'égale reconnaissance de l'engagement de toutes et de tous ?

la protection du pouvoir d'achat des professionnels des hôpitaux dans les différents secteurs. Aussi, à côté des revalorisations salariales prévues par l'accord du Ségur de la santé pour la fonction publique hospitalière, avons-nous pris des mesures en faveur du pouvoir d'achat des personnels des établissements privés

Les revalorisations des carrières et des rémunérations des sages-femmes, ainsi que la prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers et les cadres de santé, ont également été mises en place dans le privé, avec des financements associés. Par ailleurs, vous l'avez signalé, en ce qui concerne les majorations des nuits et des gardes, les mesures mises en oeuvre à la suite de la mission flash sur les urgences et les soins non programmés sont exceptionnelles et transitoires. Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, et sous l'autorité de la Première ministre, François Braun et moi-même travaillons à des systèmes de valorisation plus pérennes pour reconnaître l'engagement spécifique lié à ce travail de nuit. Nous menons également un travail en profondeur sur la permanence des soins. il nous faut mieux associer les acteurs publics et privés pour prendre en charge tous nos concitoyens, même pendant la permanence des soins. La synergie est possible. Elle l'a été pendant la crise sanitaire, nous essayons de la pérenniser.

uniquement, pour l'instant, dans le cas des majorations, les personnels non médicaux des hôpitaux publics, et non pas ceux des hôpitaux privés. Nous souhaitons que tous les personnels qui travaillent de la même façon soient reconnus.

Aujourd'hui, l'émotion est forte et la vague d'indignation nous submerge tous. Mais demain, qu'en sera-t-il ? La question du harcèlement risque de retomber dans l'oubli, pendant que des jeunes continueront de souffrir. Monsieur le ministre, je vous ai rencontré en février dernier avec ma collègue Colette Mélot. Vous sembliez alors très mobilisé

n'est pas connu dans de nombreux établissements. Les associations engagées sur ce sujet se voient refuser l'accès à certains collèges, au motif que tout va bien. Tout cela est inadmissible et ne peut plus durer ! Monsieur le ministre, avez-vous enfin l'intention de rendre obligatoire l'application des dispositifs existants ? Vous déciderez-vous à augmenter les moyens de contrôle de la mise en oeuvre effective des mesures par un renforcement des recrutements des personnels éducatifs et médico-sociaux qui manquent cruellement ? Entendez-vous renforcer la formation des enseignants et des personnels à la prévention, à la détection et au traitement du harcèlement ? Comment améliorer la coordination entre les services de l'éducation nationale, de la police et de la justice, afin que la parole de l'enfant soit prise en compte et qu'il soit et se sente protégé ?

mesure a été transmis hier au Conseil d'État. Il s'agit enfin de former massivement les personnels de l'éducation nationale et d'augmenter significativement les moyens alloués aux plateformes d'écoute 3018 et 3020.

maire de Magnières, village paisible de 400 habitants dans le Lunévillois, a été violemment agressé par dix individus après avoir tenté de mettre fin à un tapage nocturne. Malgré cette agression, profondément attaché à son mandat local, le maire, très choqué, ne démissionne pas. Je veux lui dire ici tout mon respect et lui apporter mon plein soutien. Toutefois, cette énième violence ne doit pas nous faire oublier l'incendie criminel du domicile du maire de Saint-Brevin-les-Pins ni le décès du maire de Signes

instructions de fermeté données aux parquets pour renforcer la réponse pénale ; mobilisation accrue des forces de police et de gendarmerie sur le terrain aux côtés des élus. Malgré cela,

déshumanisation de la société qui agresse nos policiers, nos pompiers et tue nos soignants, nos enseignants et nos élus ! Monsieur le garde des sceaux, quand agirez-vous pour faire appliquer concrètement des sanctions pénales exemplaires,

pour violences aggravées, outrage et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'enquête est en cours, et plusieurs individus ont déjà été interpellés.

évaluer la menace et la gravité des faits, protéger instantanément et, vous l'avez dit, sanctionner,

pratique a déjà été observée à Rio de Janeiro en 2014 et à Shanghai en 2010 lors de l'exposition universelle, avec les dérives que l'on sait. Ces déplacements choquent. Ils posent la question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes déplacées dans les régions où elles sont envoyées. des questions sur les liens entre l'État et les collectivités. En effet, il semble que les maires découvrent ces déplacements sans en avoir été informés en amont et sans que leur avis ait été sollicité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur les modalités de ces déplacements ? Comment la répartition territoriale des sans-abri franciliens est-elle réalisée ? Les élus locaux sont-ils consultés ou placés devant le fait accompli ? Quel accompagnement social est-il prévu pour les personnes déplacées ? Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que les maires ont besoin d'un peu plus de transparence et de considération ? La parole

réplique. Monsieur le ministre, je prends acte de votre réponse. Toutefois, vous comprendrez qu'après l'épisode de Saint-Brevin-les-Pins, il serait regrettable de créer de nouvelles tensions avec les maires, qui ont souvent l'impression d'être tenus pour quantité négligeable. Très bien ! Sans verser dans l'amalgame, la comparaison s'impose aussi avec la situation des migrants. Là encore, une répartition territoriale est parfois faite sans que les élus aient leur mot à dire. Les décisions de ce type, je pense que vous le comprenez, doivent être prises en concertation avec les collectivités locales, ne serait-ce que pour assurer leur succès.

l'accalmie a été de courte durée. Dans le Sud-Ouest, c'est la sidération. Depuis sept ans, chaque vague a été plus violente que la précédente. Tous les modèles ont été touchés, particulièrement l'élevage en plein air, toutes les ripostes dépassées, y compris la claustration, tous les territoires frappés et l'ensemble de la filière touchée. dernier, vous annonciez « entendre la désespérance », tout en confirmant une campagne de vaccination pour octobre prochain. Enfin ! Enfin semble se briser le tabou relatif à la vaccination aviaire. Mais octobre est un horizon lointain, extrêmement lointain, car la filière avicole, particulièrement la filière gras du Sud-Ouest, est à genoux. Beaucoup d'éleveurs ont baissé les bras. Beaucoup se sont endettés pour appliquer les mesures de biosécurité. Beaucoup attendent encore les indemnités des abattages antérieurs. antérieurs. La vaccination n'est pas la panacée, mais c'est une réponse dont on n'a que trop longtemps attendu la mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle les quatre chambres d'agriculture des départements concernés réclament pour cet été le déploiement du vaccin.

quelle sera la part à la charge des éleveurs, eux qui attendent toujours le versement des indemnisations des abattages antérieurs ? Enfin, et surtout, peut-on dans le Sud-Ouest accélérer le processus de vaccination ?

Monsieur le ministre, je comprends les problèmes techniques qui s'opposent à une vaccination rapide. Mais, dans ce cas, il faut un plan d'urgence. Sinon, quand le vaccin arrivera, les éleveurs ne seront plus là ! La parole est à M. Patrice Joly, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

la Commission européenne a dressé ce constat : « La France est caractérisée par des disparités régionales croissantes, qui vont au-delà du clivage persistant entre régions métropolitaines et ultrapériphériques. » La Commission ajoute que « la fracture entre zones urbaines et zones rurales, en termes de dynamisme économique et de perspectives de croissance, est devenue une préoccupation publique » et qu'il importe de « remédier aux déséquilibres régionaux pour, notamment, améliorer les perspectives de croissance à long terme de la France ». Enfin, la Commission préconise au Conseil de demander à la France- je reprends sa formulation -de « procéder à la mise en oeuvre rapide de programmes de politique de cohésion, en lien avec le plan de relance et de résilience », en vue d'accélérer une transition écologique, sociale, économique et numérique à la fois équitable et inclusive. Aussi, monsieur le ministre, j'aimerais entendre votre avis sur ce diagnostic impitoyable et savoir comment le Gouvernement envisage de répondre aux recommandations de la Commission. La parole est à M. le ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement.

La parole est à M. Cédric Perrin, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre des armées, même s'il est retenu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Dans quelques mois se tiendront les jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une chance, mais c'est aussi une charge d'un point de vue sécuritaire.

espérer le contraire. L'enjeu est crucial. La représentation nationale, les Français et les visiteurs du monde entier ont besoin d'être rassurés. Notre dispositif de lutte anti-drones est-il, oui ou non, opérationnel ?

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour le groupe Les Républicains. la ministre, après les déclarations successives d'un certain nombre de vos collègues, Mme la Première ministre l'a confirmé lundi dernier : le Gouvernement envisage bel et bien d'interdire l'installation et le remplacement de chaudières à gaz dans l'ensemble du parc immobilier existant, et cela dès 2026, à l'issue d'une concertation avec les acteurs de la filière. L'objectif de décarbonation de notre mix énergétique est maintenant largement admis, même si la France ne représente que 1 % des émissions de CO2 dans le monde. Il faut bien sûr trouver des solutions rapides et concrètes pour aller dans ce sens, mais certainement pas, comme le dirait le Président de la République, pour « emmerder les Français Or une telle mesure pénaliserait très lourdement les 12 millions de foyers qui se chauffent actuellement au gaz : les solutions de substitution, comme les pompes à chaleur, coûtent environ trois fois plus cher qu'une chaudière à gaz performante. cette mesure déstabiliserait une filière en pleine mutation, qui attend des marques de confiance pour continuer à promouvoir la production de biogaz sur notre sol. En réalité, notre pays a besoin d'une plus grande constance dans la parole de l'État. Il a surtout besoin d'en finir avec une politique écologique punitive, qui multiplie les interdictions.

de planifier, afin de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs que vous avez cités : d'une part, les Français qui, aujourd'hui, sont équipés de chaudières fossiles ; de l'autre, toutes les filières qui gravitent autour de ces installations.

évidemment sur les secteurs du bâtiment et du logement. Notre objectif, c'est d'avoir des logements moins énergivores et moins émetteurs de carbone. C'est une nécessité pour notre planète. C'est aussi

il ne s'agit pas de prendre des solutions drastiques et immédiates. Mais gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est anticiper. C'est ce que nous faisons, au bénéfice des Français et de nos entreprises.

Ne laissez pas les foyers les plus modestes supporter une mesure totalement déconnectée de leur réalité du quotidien. Nous en

d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, maintenant provisoirement

il y a près d'un an, dans cet hémicycle, la majorité d'entre vous était d'accord pour voter des mesures tendant à minimiser les effets d'une inflation que nous savions croissante.

qui ont été préservés de la hausse des prix qui s'en serait ensuivie. Sans ce plafonnement, l'indice de référence des loyers se serait établi à 6,26 % sur un an. Ainsi, à la faveur de cette mesure, la hausse de l'IRL a été quasiment divisée par deux.

Voilà pourquoi la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui revêt une grande importance. Oui, nous avons encore besoin de protéger nos petits commerces Nous devons les protéger en prolongeant un dispositif équilibré dans son périmètre, dans sa durée et dans son intensité. J'insiste sur ces termes,

grande anticipation des prévisions d'inflation nous plaçait inévitablement dans une situation de fragilité juridique. Il n'est jamais neutre que l'État intervienne dans les relations contractuelles privées. au travers de la proposition de loi, nous avons pris garde à cibler les commerçants les plus exposés, à savoir les TPE et les PME, c'est-à-dire les entreprises qui ont les marges les plus faibles et le moins de latitude dans leurs négociations avec les bailleurs, en particulier avec les foncières. borner cette intervention dans le temps, soit jusqu'au premier trimestre 2024, quand l'inflation, pour soutenue qu'elle demeure, devrait avoir nettement reflué. Au-delà de cette mesure rapide, ponctuelle et dictée par la nécessité, comme Olivia Grégoire a eu l'occasion de le dire aux députés la semaine dernière, nous avons lancé, voilà quelques semaines, C'est le lieu où évoquer les mutations du commerce et les thématiques structurelles qui vont bien au-delà du problème conjoncturel de l'inflation.

sujet. Le plafonnement de l'IRL doit être voté avant le 1 octobre 2023, j'y insiste. Il n'y avait donc pas d'urgence à présenter un texte. Nous voulions essayer de donner de la visibilité aux Françaises et aux Français, compte tenu du contexte actuel. C'est pour cela que nous avons proposé un texte qui pouvait être adopté avant le 30 juin 2023, même s'il n'y a pas d'obligation, puisque nous avons, je le répète, jusqu'au 1 octobre.

Plutôt que d'évaluer trop précisément, nous faisons le pari scientifique d'appliquer aux mêmes problèmes les mêmes solutions- elles ont fait leurs preuves -, à savoir la prolongation technique du dispositif déjà existant, qui a permis de limiter la hausse des loyers à 2 % en 2022.

en votant contre ce texte, vous acceptez que les locataires du parc privé encaissent une hausse de loyer de près de 10 %, alors que nous voulons tous, je le crois, préserver leur pouvoir d'achat. En 2022, un bailleur a donc pu revaloriser son loyer d'au maximum 3,6 %. En 2023, sans le vote du prolongement, un bailleur privé pourra revaloriser son loyer jusqu'à 6,1 %. Ceux qui refusent le plafonnement acceptent donc une hausse de près de 10 % des loyers pour l'année 2022-2023, soit 60 euros par mois en moyenne de plus pour les locataires du parc privé.

il aura permis 1 milliard d'euros d'économies par an pour les locataires du parc privé, qui s'ajoutent aux revalorisations structurelles décidées en 2023 pour les APL.

% dans le parc locatif social et privé. En pratique, la hausse mesurée par l'Insee a été de 2 % en 2022, contre 0,6 % en 2021.

J'ai confiance en eux. Je sais que certains sont des propriétaires modestes et qu'ils sont obligés d'augmenter les loyers pour faire face à l'inflation. Eh oui ! Je sais que, pour la majorité des autres, quand ils le peuvent, ils prennent part à l'effort de solidarité et n'augmentent pas les loyers.

Aussi, l'indice de revalorisation des loyers ne va pas s'ajuster immédiatement. La prolongation permet donc d'agir en responsabilité, en préparant au mieux un avenir encore incertain.

du texte actuel les laissent donc libres des loyers qu'ils fixeront au 1 janvier 2025, même si je sais pouvoir compter sur leur responsabilité pour limiter la hausse quand c'est nécessaire.

et quatre amendements ! ... uniquement pour faire passer un message de colère vis-à-vis de la procédure parlementaire n'est pas à la hauteur des enjeux et de la situation difficile que vivent nos concitoyens.

en urgence de cette proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par le député Thomas Cazenave. Elle a pour objet de prolonger à hauteur de 3,5 %, jusqu'au premier trimestre 2024, le plafonnement de la hausse de l'indice des loyers commerciaux et de l'indice de référence des loyers d'habitation, qui avaient été décidés, respectivement, jusqu'au premier trimestre 2023 et jusqu'au deuxième trimestre 2023, dans le projet de loi portant que nous avons voté l'été dernier. L'examen de cette proposition de loi m'amène à formuler deux séries de remarques, sur la méthode tout d'abord, sur le fond ensuite. En ce qui concerne la méthode, je fais le quintuple constat

C'est donc en janvier ou février dernier que nous aurions dû examiner un projet de loi de prolongation, et non aujourd'hui dans la précipitation. De fait, cette proposition de loi a été déposée le 23 mai. Elle a été examinée par l'Assemblée nationale moins d'une semaine plus tard en commission et en séance. Dans cette course de vitesse législative, notre commission a été contrainte de l'examiner hier, moins de sept jours après, et vingt-quatre heures seulement avant son examen en séance publique. Je voudrais rappeler que, en application de l'article 42, alinéa 3, de la Constitution, la discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt, puis, devant la seconde assemblée, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines, et qu'un délai de deux semaines est ménagé entre l'examen en commission et la séance. Les conditions d'examen de cette proposition de loi dépassent les bornes de ce qui est admissible si l'on veut mener un travail parlementaire sérieux. Dans ces délais, il est naturellement impossible d'organiser une véritable consultation des multiples parties prenantes. En effet, les différents acteurs ont été pour la plupart placés devant le fait accompli. À ma connaissance, et à la différence du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dont nous avons été saisis l'été dernier, aucune véritable concertation n'a été organisée entre les parties

En choisissant de se cacher derrière le faux-nez d'une proposition de loi, le Gouvernement se dispense en outre de toute étude d'impact. Pourtant, l'an passé, le coût pour les propriétaires du plafonnement de la hausse de l'indice de référence des loyers d'habitation avait été évalué à 705 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable de l'indice des loyers commerciaux, elle avait effectivement été plafonnée par un amendement de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne. Elle n'avait donc pas fait l'objet d'une étude d'impact, mais, à tout le moins, elle résultait d'une concertation. Enfin, en passant par une proposition de loi, le Gouvernement se dispense de prendre les indispensables mesures d'accompagnement financier et d'apporter un certain nombre de garanties aux bailleurs comme

Cet état de fait me conduit à formuler ma seconde série de remarques sur le fond du texte. La mesure de prolongation que l'on nous présente comme indispensable et urgente ne peut dispenser le Gouvernement d'une véritable politique en matière de logement et de pouvoir d'achat. Limiter la hausse des loyers face à une inflation certes élevée n'est qu'une réponse partielle et de court terme à un problème beaucoup plus large.

qui changeront la donne ! Il nous faut relancer l'investissement et l'accession de manière beaucoup plus ambitieuse. Mais comment voulez-vous encourager la location de logements contre la location saisonnière si vous faites passer le message que les indices de références ne seront pas respectés, alors que les loyers saisonniers, eux, ne sont pas régulés De plus, les charges pesant sur les propriétaires ne sont pas allégées. La revalorisation des valeurs locatives sur l'inflation pour le calcul de la taxe foncière n'a pas été plafonnée. L'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) la chiffre à près de 3 milliards d'euros. N'oublions pas non plus que la rénovation énergétique des logements est à la charge des propriétaires. Le plafonnement n'est pas moins lourd de conséquences pour les bailleurs sociaux. En effet, l'inflation se répercute notamment sur leurs emprunts à long terme,

de 0,5 % à 3 % en un an, les charges d'intérêts des organismes de logement social se trouvent alourdies de 3,75 milliards d'euros, ce qui affecte très fortement leur capacité à investir. Or cette hausse se répercute également sur l'IRL, donc les loyers, mais également sur les APL et les salaires. En bloquant ce mécanisme sans compensation, le Gouvernement impose une nouvelle ponction aux bailleurs sociaux, alors que la réduction de loyer de solidarité (RLS) représente déjà 1,3 milliard d'euros par an. Comment espérer ensuite qu'ils puissent répondre présents aussi bien en matière de rénovation que de construction ? En prolongeant le plafonnement de la hausse des loyers, le Gouvernement n'apporte en outre qu'une réponse partielle à la baisse du pouvoir d'achat. Comme je l'ai déjà indiqué, ce texte n'offre aucune garantie sur la revalorisation des aides personnelles au logement en faveur des locataires les plus modestes. Au cours des années passées, la hausse des APL a été déconnectée de l'IRL. L'exemple le plus flagrant est est le forfait de charges, dont l'augmentation a été deux fois moins rapide que la dépense réelle au cours des dernières années. D'ailleurs, il ne couvre plus que 40 % des charges effectives. Or, nous le savons tous ici, les charges augmentent plus vite que les loyers ! Enfin, la limitation de la hausse des loyers n'exonère pas le Gouvernement d'une réflexion sur la hausse des salaires. C'est tout particulièrement flagrant dans les commerces qui sont confrontés à une situation difficile : la fréquentation des commerces non alimentaires aurait reculé de 20 %. Selon les chiffres publiés en avril dernier par l'Insee, les achats alimentaires ont diminué de 10 % en un an, et la baisse est beaucoup plus importante sur certaines catégories de produits. Limiter la hausse des loyers ne permettra pas de redonner vraiment du pouvoir d'achat à certains Français, mais elle en prendra à d'autres : les propriétaires. C'est pour l'ensemble de ces raisons que la commission des affaires économiques a décidé de rejeter cette proposition de loi.

Ils ne peuvent pas absorber une baisse de la rémunération des loyers et une hausse du taux du livret A : il leur faut une compensation ! Par ailleurs, nous considérons que le sujet du prix du logement est essentiel. Sur ce point, je ne comprends pas la position de la majorité relative présidentielle

au coeur de l'été 2022, le Gouvernement avait mis à l'ordre du jour des débats parlementaires un projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette démarche était opportune et très attendue par les Français, qui étaient confrontés à une inflation généralisée.

de la variation annuelle de l'indice des loyers des petits commerces, issu, entre autres, d'un amendement de mon groupe. L'article 12 prévoit, quant à lui, le plafonnement de l'indice de référence des loyers au profit des ménages. Concrètement, la revalorisation n'a pu excéder 3,5 %, pour protéger les locataires, ainsi que les petits propriétaires, qui subissent également une hausse de leurs charges. Naturellement, le gel des loyers commerciaux et locatifs aurait sans doute été préférable- le loyer représentant le plus gros poste de dépenses des ménages,

20 % sur un an. Le constat des acteurs du logement est sans appel : 4,1 millions de personnes sont sans logement ou mal logées ; 12,1 millions de Français sont fragilisés par la crise du logement ; 12 millions de nos compatriotes souffrent de précarité énergétique ; 2,3 millions de ménages sont en attente d'un logement social.

Le Gouvernement a classé ses différentes mesures selon cinq axes : favoriser l'accession à la propriété ; favoriser l'accès à la location ; soutenir la production et la rénovation des logements sociaux ; relancer la production de logements ; enfin, amplifier la rénovation énergétique et thermique des logements du parc privé.

comme la volonté de « lever les freins juridiques à la production de logements compatibles avec nos objectifs de sobriété foncière » : le célèbre « en même temps

et résilience ? ... Voilà des années que les acteurs du secteur nous alertent sur leurs difficultés croissantes. Résoudre la crise du logement, c'est notamment redonner des marges de manoeuvre sur le terrain, ainsi que du pouvoir d'achat aux Français. nous avons la responsabilité d'agir avec raison, et non à la va-vite. C'est pourquoi nous sommes nombreux à dénoncer la méthode et l'approche retenues pour cette proposition de loi. Déposé il y a seulement deux deux semaines, voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière et transmis au Sénat dans la foulée, ce texte a un goût de frustration. Pis, il donne un sentiment de panique à bord.

À défaut d'une politique plus ambitieuse, la majorité présidentielle se contente de reconduire, dans l'urgence, un dispositif théoriquement temporaire. Comme lors de l'examen en commission hier matin, le RDSE s'opposera à la motion tendant

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Oui, les conditions d'examen de cette proposition de loi manifestent un mépris du Parlement en général et du Sénat en particulier. L'urgence décrétée pour examiner ce texte en deux semaines ne s'explique que par l'impréparation du Gouvernement. Mais peut-être est-elle le fruit de désaccords plus profonds

Le Gouvernement prend le Sénat pour une chambre d'enregistrement. Où est l'étude d'impact ? Nulle part. Où est l'évaluation des mesures prises l'été dernier ? Nulle part. Nulle part. De combien les loyers et les valeurs locatives commerciales ont-ils effectivement augmenté ? Mystère. Quels sont les coûts et les conséquences pour les propriétaires privés et pour les bailleurs sociaux ? Aucune idée. Mes chers collègues, on nous demande aujourd'hui de voter non seulement à la sauvette, mais aussi à l'aveuglette Ce texte manifeste également une forme de mépris à l'égard du secteur du logement et de tous ses acteurs. Il n'a fait l'objet d'aucune concertation, et la plupart des acteurs ont été mis devant le fait accompli. Mais après tout, quoi de surprenant,

Prolonger le plafonnement des indices locatifs en urgence ne fait pas une politique du logement construite et cohérente de long terme. Le discours de la Première ministre lundi soir a montré que le Gouvernement prenait la crise du logement à la légère ; je le dis avec gravité. Tel est, monsieur le ministre, le taux d'augmentation du nombre de demandeurs de logements sociaux depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Voilà le résultat de la politique du logement conduite depuis 2017. Le CNR Logement est un véritable rendez-vous manqué. De l'avis général, ses conclusions témoignent d'une incompréhension totale des investisseurs, publics ou privés, petits et grands, trop taxés, sans visibilité, sans stabilité, sans respect des engagements ; des entreprises, qui s'inquiètent à juste titre du devenir d'Action Logement pour leurs salariés ; des élus locaux, auxquels on ne donne plus les moyens d'accueillir les nouveaux habitants

Pourtant, des mesures structurelles pour relancer la construction et débloquer le parcours résidentiel étaient possibles. Je pense par exemple au soutien aux maires bâtisseurs. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, les maires n'ont plus de recettes fiscales dynamiques et pérennes leur garantissant une augmentation de leurs ressources, en lien avec la avec la croissance de la population et les constructions nouvelles. Et vous vous étonnez qu'ils soient plus frileux à construire ! Il est nécessaire d'aller bien au-delà d'une prime au permis ou d'une compensation partielle et temporaire

devons leur rendre le pouvoir d'attribution des logements sociaux, car nos maires n'en peuvent plus de devoir construire sous contrainte et de ne pas pouvoir donner satisfaction à leurs propres administrés Autre piste que vous auriez pu explorer : la suppression de tout ou partie de la réduction de loyer de solidarité, qui pèse 1,3 milliard d'euros par an sur les capacités d'investissement des bailleurs sociaux,

Enfin, vous auriez pu débloquer le parcours résidentiel, plus particulièrement l'accès à la propriété, ce fameux « rêve français », qui n'est peut-être pas le vôtre, mais qui est légitime pour des milliers de nos compatriotes. Leur dénier ce droit revient à les condamner à une forme de déclassement. Quant au pouvoir d'achat, ainsi que l'a dit Mme le rapporteur, à la différence du texte voté l'année dernière, vous n'offrez aucune garantie pour les plus modestes. Quelle sera l'augmentation des APL dans le prochain projet de loi de finances (PLF) ? Quelle sera l'augmentation du forfait pour charges ? Mystère. En rejetant ce texte et en soutenant la question préalable déposée par la commission, le groupe Les Républicains ne souhaite pas s'opposer à une solution pour nos concitoyens et nos PME, solution qui sera vraisemblablement adoptée à l'Assemblée nationale. Monsieur le crier notre colère avec force et conviction et dire notre totale opposition à l'ensemble de la politique du logement méticuleusement déconstruite depuis 2017. Ce texte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

il y a un peu moins d'un an, le 29 juillet dernier, dans cet hémicycle, nous adoptions le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Il s'agissait de protéger les Français, ménages et professionnels, face au choc inflationniste qui frappait notre pays. Parmi les différentes mesures adoptées, l'une d'entre elles consistait à plafonner à 3,5 la revalorisation annuelle des indices locatifs, dits « IRL » pour les particuliers et « ILC » pour les commerçants. Pourquoi avoir attendu le début du mois de juin pour proposer la prorogation d'un dispositif qui arrivera à son terme à la fin du mois ? On peut tout de même se poser la question, même si, je l'admets, ce n'est pas vraiment ce qui doit nous préoccuper cet après-midi. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'objet de cette proposition de loi, qui vise à prolonger d'une année, soit jusqu'au premier trimestre 2024, le dispositif de plafonnement à 3,5 % des indices locatifs dans l'Hexagone et à 2,5 % outre-mer. Rappelons que, sans ce dispositif, cette revalorisation serait aujourd'hui de plus de 6 %.

au supermarché, à la pompe à essence ou à celle de l'énergie reste difficilement surmontable pour les ménages les plus fragiles. Ils diront aussi que certains petits commerçants et artisans ne pourront faire face à une hausse de leur loyer qui viendra se conjuguer à celle de l'énergie, des matières premières et à la baisse des commandes. En cela, ils auront raison : beaucoup sont de fait déjà pris à la gorge, avant même toute éventuelle revalorisation du montant de leur loyer. loyer. Faudrait-il ne rien faire et laisser les loyers exploser pour noyer complètement ceux qui parvenaient tout juste à maintenir la tête hors de l'eau ? Bien sûr que non ! Geler totalement les loyers et pénaliser l'intégralité des propriétaires ? Non

parmi les locataires, il y a aussi le jeune couple qui ne veut pas, ou ne peut pas, contracter un prêt immobilier. Il faut le dire, sans provocation : tous les locataires ne sont pas à plaindre et tous les propriétaires ne sont pas à envier. Évitons les caricatures qui opposent le locataire pauvre au propriétaire nanti, car, dans chacune de ces deux catégories, certains éprouvent exactement les mêmes difficultés à régler leurs charges à la fin du mois, voire bien plus tôt. Certains propriétaires, comme certains locataires ou certains commerçants, font face à une augmentation des charges de copropriété, de la taxe foncière et des travaux de rénovation énergétique dont beaucoup devront s'acquitter et que les aides de l'État ne couvrent pas intégralement. Cette proposition de loi nous semble ainsi être une mesure d'équilibre, d'effort réparti : elle protège les ménages et les commerçants d'une hausse brutale de leur loyer, sans pénaliser lourdement les propriétaires.

S'il peut représenter une solution de court terme, voire de moyen terme en l'espèce, visant à contenir la spirale inflationniste et à préserver le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas vocation à perdurer au-delà de 2024,

La France connaît des problèmes structurels de logement, sur lesquels l'ensemble des acteurs, constructeurs, promoteurs, bailleurs et collectivités locales alertent depuis des années. Il faudrait construire entre 400 000 et 500 000 logements par an. Force est de constater que le compte n'y est pas. Le Gouvernement partage ce constat : il a dévoilé ce lundi un plan contre la crise du logement. Les difficultés se sont nettement aggravées depuis la hausse des coûts des matériaux et celles des taux d'intérêt, qui rendent de plus en plus difficile l'accès au crédit immobilier pour nombre de Français.

d'opinion publique (Ifop) nous apprend qu'une fois les dépenses essentielles réglées, 31 % des Français se retrouvent avec moins de 100 euros sur leur compte dès le 10 du mois. plus, de nombreux locataires ne parviennent plus à payer leur loyer dans les temps : selon l'Union sociale pour l'habitat (USH), les retards de paiement de plus de trois mois ont augmenté de 10 % en 2022.

précaires. Bien sûr, ce plafond a le mérite d'exister face aux 6 %, 8 % ou 10 % de hausse que l'on nous prédit si ce texte n'était pas adopté. Mais le problème ne vient pas uniquement de l'inflation : il est bien plus profond. On notait, à la fin de 2022, une hausse de plus de 7 % des demandeurs de logements sociaux, alors même que leur production a atteint un nouveau record à la baisse de 95 000 constructions en 2022, le niveau le plus bas depuis quinze

Alors que nous demandons des efforts importants, notamment en matière de rénovation énergétique, s'attaquer aux dépenses d'investissement, c'est mettre à mal toute la politique du logement Face à ces problèmes de construction et d'aggravation de la précarité des ménages, il est de notre devoir d'aider au mieux les locataires, en abaissant le plafonnement de la hausse des indices locatifs. Alors que les locataires ont déjà subi une hausse de 3,5 % l'an dernier, ils pourraient connaître une nouvelle hausse équivalente si ce dispositif était adopté. C'est pourquoi nous proposons de fixer le plafonnement à 1 %, ce qui permettrait de protéger les locataires en compensant quelque peu l'inflation pour les propriétaires, sachant que l'augmentation des charges locatives pèse totalement sur les locataires. Encore une fois, ce bouclier de loyer ne résoudra pas la crise, qui, bien qu'elle soit aggravée par le contexte actuel, est profondément structurelle. Il y a tout d'abord un véritable problème dans la méthode de calcul des indices locatifs.

face à l'inflation qui combine les effets de la sortie de la crise sanitaire et le bouleversement géopolitique de la guerre en Ukraine, nous avons fait le choix, parmi une batterie de mesures visant à protéger les Français,

Madame le rapporteur, hier, en commission, vous avez déploré l'impossibilité d'organiser un cycle d'auditions compte tenu des délais. Je le regrette également, car cela nuit à la qualité des travaux de notre assemblée, d'autant plus que vous avez eu l'amabilité de bien vouloir reprendre les travaux en cours.

Le Parlement doit prendre le temps nécessaire pour mieux légiférer. Le temps parlementaire n'est pas accessoire et, à l'avenir, nous souhaitons une meilleure anticipation des mesures législatives provisoires. Cela étant, le Sénat est capable, grâce à ses exceptionnels fonctionnaires, de légiférer dans l'urgence quand la situation l'exige. Les deux articles de ce texte de loi sont facilement compréhensibles

Les estimations montrent que l'ILC et l'IRL resteront à un niveau élevé, probablement autour de 6 % en glissement annuel, pour atteindre progressivement 3,5 % au deuxième trimestre de l'année 2024. Dès le mois de juillet 2023, la croissance de 6 % des loyers des locataires, des TPE et des PME est possible. Mes chers collègues, je sais que la majorité sénatoriale n'est pas le parti de la pressurisation des Français.

Ce texte étant présenté dans des délais très contraints, la concertation n'a pu être menée, et nous le regrettons. Mais rejeter le texte, même pour des motifs de forme compréhensibles, ce serait laisser penser que nous serions prêts à laisser les Français et les

provoquée par des événements exogènes aux cycles économiques naturels. Le Président de la République a promis de tout mettre en oeuvre pour protéger les plus faibles dans la tempête que le monde traverse depuis la crise de la covid-19 et la guerre en Ukraine. C'est notre ligne. Pour ces raisons, le groupe RDPI votera contre la question préalable et réaffirme son soutien plein et entier à cette proposition de loi qui protège les locataires et les commerçants. Mes chers collègues, je vous invite à la voter conforme.

alors que leur capacité d'action est déjà entravée par la multiplication par plus de trois des taux d'emprunt, indexés sur la rémunération du livret A, ainsi que par la diminution du loyer de solidarité, qui représente pour eux une perte annuelle de 1,3 milliard d'euros.

pénalise surtout les locataires en situation d'impayés de loyer, en les menaçant d'une amende de 7 500 euros et en accélérant les procédures d'expulsion. Monsieur le ministre, j'attire tout particulièrement votre attention sur la situation des habitants des quartiers prioritaires En 2022, la moitié des organismes HLM a enregistré une augmentation de plus de 10 % du nombre de loyers en retard de paiement de plus de trois mois. Cette tendance va se confirmer en 2023. Les élus et les associations attendent de l'État un véritable plan d'urgence répondant aux enjeux économiques, écologiques et sociaux des quartiers populaires. Traiter la question du logement

de ménages en difficulté financière en décembre 2022. Cette tendance préoccupante est largement liée à l'explosion des factures de gaz et d'électricité, qui s'ajoutent aux loyers.

ces mesures s'imposent à l'État. Elles répondent aux besoins d'investissement comme à la problématique des ménages en difficulté, sans pour autant reporter le problème sur les propriétaires, notamment les plus petits d'entre eux, qui sont souvent des retraités dépendants de ce complément de revenus.

ajoute l'engagement de la procédure accélérée, qui impose un examen du texte dans l'extrême urgence : il ne nous a été laissé qu'une semaine pour élaborer un rapport et une journée seulement sépare l'examen du texte en commission de son passage en séance publique

et ruraux », dresse un constat alarmant du bilan du Gouvernement en matière de logement et souligne que les dispositifs de régulation du marché immobilier en place incitent les investisseurs à privilégier la plus-value, plutôt que la rentabilité locative raisonnable basée sur les loyers. Cela rend le marché immobilier privé encore plus spéculatif. À la fois en raison de la méthode employée, de nos réserves envers le dispositif proposé, qui charge les propriétaires de la responsabilité de l'inflation, alors même que la protection du pouvoir d'achat en matière alimentaire est insuffisante, et de l'absence de mesures visant réellement à remédier à la crise du logement,

L'envers du décor, c'est le Président de la République qui qualifie la politique du logement de notre pays de « système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective Comme à votre habitude, vous prétendez partager les constats et être conscient de l'ampleur de la crise. Et quelle crise, monsieur le ministre : 2,4 millions de personnes attendent aujourd'hui un logement social et 330 000 personnes restent sans domicile.

qu'ils sont les mieux placés pour relancer la dynamique de construction perdue depuis 2017, vous leur envoyez des signaux négatifs. Il est grand temps de leur redonner confiance, plutôt que de les ignorer.

après la discussion générale, afin de ne pas limiter l'expression des groupes politiques. Chacun a pu ainsi donner son opinion, avancer ses propositions

dans des délais complètement anormaux. Cette fausse urgence sert à cacher l'impréparation du Gouvernement sur ce sujet, alors que les délais sont connus depuis un an.

Il n'y a pas eu de concertation, non plus que d'évaluation. Comme je l'ai indiqué, nous ne sommes pas hostiles par principe à des mesures d'urgence, quand celles-ci se justifient ; nous les avons d'ailleurs votées l'an passé. Alors, les

comme un signe de mépris par l'ensemble des acteurs du secteur du logement, qui ont travaillé pendant sept mois pour presque rien. La construction traverse une crise très grave. Le nombre de réservations auprès des promoteurs est tombé au niveau du printemps 2020, au coeur de la crise sanitaire- c'est dire l'importance du marasme. La RLS, la réduction de loyer de solidarité, et la hausse du taux du livret A assèchent les capacités de construire et de rénover des bailleurs sociaux, alors que le nombre de demandeurs a franchi la barre des 2,4 millions. Hier, devant la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, que je préside, Christophe Béchu indiquait

90 % des communes qui ne sont pas situées en zone tendue. Les demandeurs de logements sociaux n'ont jamais été plus nombreux, mais on continue d'étrangler les bailleurs sociaux, qui seraient des dodus dormants. On veut des investisseurs dans le logement locatif intermédiaire ; pourtant, face à l'inflation, on ne bloque que leurs revenus ! La France serait un paradis fiscal pour investisseurs immobiliers, selon Emmanuel Macron ; drôle de paradis que celui dans lequel, pour 38 milliards d'euros de dépenses, l'État récupère 90 milliards d'euros Depuis 2017, la stratégie du Gouvernement se résume à deux chiffres : 18 % de demandeurs de logements sociaux en plus et 81 % de recettes budgétaires nettes en plus sur le logement. Aujourd'hui, dans le domaine du logement, le dodu dormant, c'est le Gouvernement Tout cela a un impact direct sur les Français, qui peinent de plus en plus à se loger ou qui subissent des coûts prohibitifs. Le parcours résidentiel, symbole d'ascension sociale, est bloqué. Les Français se sentent déclassés

du pouvoir d'achat tout court. Mes chers collègues, telles sont les raisons qui nous conduisent aujourd'hui à proposer au Sénat d'adopter cette motion tendant de marquer clairement notre opposition à cette législation à la sauvette et à une politique du logement sans vision et sans stratégie, faite seulement de mesurettes. Y a-t-il

Les échéances étaient connues. Il incombait donc au Gouvernement d'anticiper la fin du plafonnement des loyers voté l'été dernier dans un rare consensus politique. Le texte qui nous est soumis est une insulte au travail du Parlement.

Légiférer dans l'urgence, par des mesures de blocage, n'apporte aucune solution pérenne et efficace. Nous ne pouvons donc qu'exprimer notre mécontentement en votant cette motion et en renvoyant le Gouvernement à ses responsabilités. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, explication de vote.

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je maintiens les propos que j'ai tenus lors de la discussion générale : la méthode employée par le Gouvernement pour traiter d'un sujet aussi important que l'encadrement de la hausse des loyers n'est pas acceptable.

par la diminution des dépenses des ménages causée par l'inflation. L'augmentation de l'ILC a déjà eu pour conséquence désastreuse la fermeture de nombreux magasins qui n'ont pas réussi à suivre la hausse généralisée des prix.

ou une augmentation beaucoup plus faible de celui-ci. Si les commerçants peuvent rencontrer des difficultés- je ne le nie pas -, les propriétaires sont eux aussi confrontés à la hausse de leurs charges, ne serait-ce que la revalorisation des valeurs locatives sur la base de l'inflation, qui, elle, n'est pas plafonnée.

ainsi qu'une hausse de 10 % des factures d'énergie impayées. Au sein de la catégorie durement touchée des dépenses dites « essentielles », le loyer n'est pas épargné. Le plafonnement en vigueur a certes permis de limiter la hausse à 25 euros par mois en moyenne, mais cette mesure ne suffit pas.

des APL et du forfait pour charges. Néanmoins, la décision de plafonner la hausse de l'IRL à 3,5 % est le fruit d'une volonté de compromis et de partage équilibré des charges entre propriétaires et locataires,

quand la formule pour calculer le prix du bail date de 1986 ... La révision de 2008 n'a pas porté sur les éléments qui auraient pu légitimer l'IRL, ce dernier ne tenant toujours pas compte des disparités géographiques qui existent entre la capitale, les territoires ruraux ou littoraux, les grandes et petites

de maîtriser les hausses, dans une période où l'inflation était très élevée, et de trouver une solution équitable après l'extinction du régime issu de la loi de 1948. Ce choix s'est toutefois révélé imparfait, car lorsque l'indice encadrement était défavorable à l'investissement locatif, alors que, lorsque l'indice était dynamique en raison du coût des matières premières, les loyers pouvaient augmenter plus rapidement que l'inflation.

avec un certain décalage et en la lissant. On a en effet considéré que l'inflation, ou plus précisément l'indice des prix à la consommation hors tabac et loyers, était l'indicateur le plus large

de mener une réflexion stratégique sur l'évolution des loyers, à la fois pour préserver le pouvoir d'achat des locataires et pour rendre crédible l'investissement locatif privé.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

Cet article traite d'enjeux aussi divers que les perquisitions de nuit dans le cadre des enquêtes de flagrance pour les crimes contre des personnes, le recours à la vidéotransmission pour les examens médicaux pendant la garde à vue, le renforcement du statut de témoin assisté, le recours au placement en détention provisoire préalable

Regroupées dans un seul article sans véritable cohérence, les dispositions sont difficiles à étudier et portent souvent à confusion, loin de la clarification que vous appelez En matière de procédure pénale, nous avons besoin de cohérence et de stabilité. Cet article, où se juxtaposent des mesures très techniques et des dispositions très sensibles, a du mal à y contribuer.

Il s'agit de trouver un équilibre entre efficacité des enquêtes et renforcement des droits des personnes faisant l'objet d'une perquisition. Pour ce faire, nous proposons que l'avocat puisse être présent lors des perquisitions : l'officier de police judiciaire ou le magistrat ne pourraient pas s'opposer à sa présence à son arrivée sur les lieux, même si la perquisition est déjà en cours. cours. Si la personne est suspecte et si une audition est prévue pendant la perquisition, elle doit être informée de son droit d'être assistée par un avocat, conformément aux règles sur l'audition libre ou la garde à vue.

que le droit actuel offrait déjà des garanties suffisantes, puisque, en cas d'audition au cours de la perquisition, la personne doit déjà pouvoir, à peine de nullité, être assistée par un avocat,

Il est à craindre une généralisation, voire une banalisation d'une mesure de procédure pénale dite pourtant « d'exception ». Quelles seront les garanties procédurales qui permettront d'empêcher les abus de pouvoir de la police ? Les services d'enquête bénéficient pourtant déjà de larges moyens d'intervention. Nécessité et proportionnalité sont de rigueur, surtout quand il s'agit de porter atteinte aux libertés individuelles. Si le juge d'instruction autorise de manière anticipée une perquisition de nuit dans un lieu d'habitation en raison d'un risque prévisible de dépérissement des preuves, la présence d'un avocat devra être obligatoire et systématique.

préliminaire. Cette nouvelle extension des perquisitions de nuit à des crimes de droit commun, certes en cas d'atteinte aux personnes, vient mettre à mal, comme l'a souligné ma collègue Esther Benbassa, l'équilibre entre les différents principes à valeur constitutionnelle, faisant reculer encore le principe d'inviolabilité du domicile et, ainsi, la protection attachée au domicile. Je rappelle aussi que les services d'enquête disposent déjà de nombreux moyens d'intervention, de jour comme de nuit, comme les surveillances, les dispositifs de sécurisation, les filatures et les interpellations, et qu'ils peuvent déjà pénétrer dans les domiciles en cas de réclamation de l'intérieur.

Nous sommes en effet toujours attentifs à l'affaiblissement des prérogatives du juge des libertés et de la détention ou à sa surcharge de travail, qui rend impossible l'exercice de sa mission. Nous pensons que le texte est trop déséquilibré en termes de contrôle par l'autorité judiciaire du respect des droits des personnes.

de M. le président du Parlement de Géorgie, M. Shalva Papuashvili, et d'une délégation de députés géorgiens. Après avoir été accueillie aujourd'hui à l'Assemblée vient de s'entretenir avec M. le président du Sénat. Elle est notamment accompagnée par nos collègues Alain Houpert, président du groupe d'amitié France-Caucase, et Philippe Tabarot, président délégué pour la Géorgie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires réguliers entre nos deux assemblées. Elle porte en particulier sur l'actualité internationale et européenne, dans le contexte à la fois de la guerre en Ukraine et du souhait de la Géorgie d'accéder au statut de « pays candidat À ce titre, la délégation s'entretiendra demain avec notre collègue Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Permettez-moi de souhaiter à nos amis géorgiens un séjour et des échanges fructueux, en formulant le voeu que cette rencontre interparlementaire contribue à renforcer encore nos liens d'amitié. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français.

Cette lacune peut compromettre leur droit à une défense adéquate et équitable. En instaurant une convocation écrite, nous souhaitons garantir une meilleure compréhension des droits aux personnes auditionnées. La notification écrite permettra d'expliciter clairement les droits qui leur sont accordés, y compris y compris le droit d'être assisté par un avocat lors de l'audition libre. Les auditions seront ainsi transparentes et équitables. Quel

une consultation médicale physique est obligatoire. Les personnes interpellées se trouvent parfois en état de choc et d'angoisse. Le médecin reste alors la seule personne rassurante et objective dans un milieu hostile : l'enceinte d'un commissariat. La consultation médicale physique a alors toute son importance, puisqu'elle permet de dresser un constat réel de l'état du gardé à vue. à vue. La téléconsultation médicale risque de compromettre la confidentialité des échanges entre le gardé à vue et le médecin. Il y a de sérieuses interrogations quant à la protection des données. Quelles sont alors les garanties pour protéger le gardé à vue ?

il n'en demeure pas moins que, souvent, la disposition des locaux de garde à vue ne permet pas d'assurer de manière concrète et efficace cette confidentialité dans le cadre d'une visioconférence. De même, la nécessaire autorisation du procureur de la République pour recourir à la téléconsultation ne constitue pas une garantie suffisante, dans la mesure où la décision sera prise sans que le magistrat ait vu la personne privée de liberté. La pénurie de médecins ne doit pas être contournée ou instrumentalisée aux dépens des droits des plus fragiles.

que la téléconsultation ne concerne que les majeurs non protégés. Encore heureux ! Certes, mais encore faut-il le dire ! La téléconsultation doit être mise en place avec l'accord du procureur de la République.

ou par un membre de sa famille, le recours à la téléconsultation doit être expressément accepté par celui qui sollicite l'examen. Il n'est pas imposé.

Nous comprenons bien l'intérêt d'un tel dispositif, dans la mesure où l'examen à distance permet en effet d'alléger et d'accélérer les procédures, mais nous croyons également que le rôle du médecin est trop important pour que ces procédures fassent l'objet de mesures d'allégement.

Le présent amendement vise à rendre cette possibilité systématique et obligatoire. En effet, la présence de l'avocat dès la première audition est indispensable et contribuera au renforcement des droits de la défense. La présence d'un avocat permet un équilibre des pouvoirs entre le suspect et les enquêteurs. Au cours des auditions, la personne gardée à vue peut faire face à des intimidations. Il n'est pas rare d'entendre des prévenus témoigner que des agents de police les ont dissuadés d'appeler leur avocat pour la première audition. De telles méthodes ne sont pas acceptables. L'avocat est une garantie que, dès le début de la garde à vue, les droits du gardé

tout de même bien le moins que le suspect soit mieux informé que tel ou tel journaliste ayant bénéficié d'une violation du secret de l'enquête, d'autant que certains organes

Mais il nous faut prendre en considération la difficulté que les délais posent. Même si nous ne reviendrons pas sur le principe, ces délais étant trop importants pour notre droit, nous nous nous adaptons et nous permettons en échange, si j'ose dire, un accès total au contradictoire pour que le suspect puisse enfin faire valoir complètement les droits qui sont les siens.

à comprendre votre amendement complexe, dont l'exposé des motifs n'était pas tellement plus éclairant. Nous voyons que vous

indépendamment des exemples qui ont pu être donnés. Elles ne donnent pas toujours lieu à des articles dans la presse ou à un feuilleton. En tout état de cause, nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont on pourrait permettre un exercice du contradictoire au cours de ces enquêtes préliminaires. En réalité, c'est un peu la quadrature du cercle. Évidemment, la proposition de prolongation du délai n'est pas plaisante.

n'est pas conforme à ce que vous nous avez présenté, du moins nous semble-t-il. Le point de départ du contradictoire tel que vous nous l'avez expliqué voilà quelques secondes ne correspond pas à ce que nous lisons. Je pense que les rapporteurs ont raison de vous mettre

que les données de l'étude d'impact étaient inexactes et que vous avez pu voir à l'expérience que les stocks de procès-verbaux (PV) dans les commissariats et les gendarmeries étaient beaucoup plus importants et anciens que vous ne l'aviez pensé initialement. D'où votre pragmatisme actuel. La

souhaitons autoriser le mis en cause et son avocat à demander la nullité d'actes devant le juge des libertés et de la détention, avec une possibilité d'appel devant la chambre de l'instruction. actuelle, il existe finalement peu de moments où le contradictoire est possible dans les enquêtes préliminaires, ce qui désavantage à nos yeux les droits de la défense. Quel est l'avis de la commission Mme la rapporteure évoquent la possibilité d'avoir accès à un dossier expurgé. Nous pensons que l'article 61-1 du code de procédure pénale contient déjà des garanties suffisantes puisque la personne est déjà informée « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ». Cet accès à un dossier expurgé viendrait alourdir la procédure et ne nous semble pas utile

là encore, à renforcer les droits de la défense et le principe du contradictoire dans les enquêtes préliminaires en permettant l'accès au dossier au plaignant et à son avocat après un délai de six mois. Actuellement, l'absence d'accès au dossier entrave la construction d'une défense solide et compromet le principe du contradictoire, ainsi que le droit à une défense équitable. Il est difficilement justifiable que l'avocat n'ait accès au dossier de son client que plusieurs années après le début de l'enquête, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre amendement a donc pour objet d'autoriser l'accès au dossier après un délai de six mois à compter du début de l'enquête préliminaire. L'avocat du plaignant pourra obtenir une copie du dossier et la transmettre à son client sous réserve, bien évidemment, de l'autorisation préalable du procureur de la République.

pour préparer leur contestation et exercer pleinement leur droit de défense. Nous ne pouvons pas le nier, la mise en examen est une étape cruciale dans une procédure pénale, au regard des conséquences qu'elle peut avoir sur la personne concernée. Nous considérons donc qu'il est essentiel de garantir un délai raisonnable pour préparer une défense adéquate. En allongeant le délai de contestation à dix jours, cet amendement tend à favoriser le respect des droits de la défense. Nous proposons

? Je pense que ces deux amendements sont excellents ! Le futur mis en examen qui sort de garde à vue n'a pas une connaissance intégrale de son dossier. Certes, son avocat a pu lui communiquer avant la mise en examen un certain nombre d'éléments.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement, qui est issu d'une recommandation du Conseil national des barreaux, vise à instaurer l'information de la partie civile lors d'une demande de « démise » en examen. Le principe du contradictoire doit être intégré au sein de la procédure de démise en examen, afin que la partie civile puisse former des observations en défense, avant la décision du juge d'instruction. Il est donc nécessaire de prévoir que la demande de démise en examen soit communiquée par le juge et la partie civile plaignante.

toutes les parties concernées lorsqu'il accède à une demande d'audition émanant d'une partie, qu'il s'agisse d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen. À l'heure actuelle, il n'est pas obligatoire pour le juge d'instruction d'informer les autres parties, qui n'ont pas le droit

compréhension de l'avancement de l'enquête et pourront pleinement exercer leurs droits à la défense. Il s'agit finalement de garantir un peu plus de transparence dans la procédure judiciaire. Quel est l'avis de la commission ? Une telle

d'une plainte simple et que celui-ci soit a rejeté sa plainte, soit n'a pas répondu dans un délai de trois mois. Un tel dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d'une victime et retarde l'entrée en action du juge d'instruction. Un certain nombre d'acteurs de la justice nous ont alertés sur cette difficulté, que nous souhaitons faire disparaître. Cet amendement vise donc à supprimer la condition de recevabilité et à revenir au système antérieur à la loi de 2007.

à Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à garantir la notification des réquisitions de non informer et de non-lieu à la partie civile, ainsi qu'à instaurer l'établissement d'un délai pour que le juge d'instruction rende son ordonnance à la suite des réquisitions du ministère public. Il est primordial d'assurer l'équité et la transparence dans la procédure pénale. La partie civile a le droit de connaître les réquisitions du procureur, qui peuvent influencer sa réparation et avoir des implications importantes sur l'issue de l'affaire. En lui accordant la possibilité de prendre connaissance de ces réquisitions et de présenter des observations à leur sujet, nous renforçons le principe du contradictoire et préservons ainsi les droits de la partie civile. Nous considérons que l'introduction d'un délai pour la prise de décision par le juge d'instruction est essentielle pour assurer l'efficacité de la procédure. En l'absence d'un tel délai, il peut y avoir des retards injustifiés dans le déroulement de l'information. Un délai clair et raisonnable permettra d'éviter les blocages et d'assurer une gestion efficace des réquisitions du ministère public, tout en préservant les droits des parties impliquées.

personnes : meurtres, assassinats, enlèvements et séquestrations, etc. À l'instar des perquisitions de nuit réalisées dans le cadre d'une enquête de flagrance, ces perquisitions de nuit ne pourraient être autorisées que dans trois hypothèses soit la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique ; soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis ; soit la perquisition est nécessaire pour permettre l'interpellation de l'auteur du crime.

amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat. En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or son intervention n'est pas prévue en cas d'écoute téléphonique sur la ligne d'un avocat sur le fondement de l'article 100 Il est donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d'un avocat, de la même façon qu'il peut déjà s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d'un avocat.

à l'activation de téléphones portables. Nous nous faisons ici le relais des avocats, qui s'inquiètent d'un tel dispositif, susceptible de porter atteinte à la confidentialité de leurs relations avec leurs clients. Cet amendement a pour objet d'interdire l'enregistrement des conversations entre un avocat et son client. 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l'exercice des droits de la défense, il serait néanmoins possible d'écouter et d'enregistrer ces mêmes correspondances. De telles telles dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l'avocat et aux droits de la défense. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'interdire explicitement l'interception et l'enregistrement des échanges entre un avocat et son client dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. La parole est à M.

l'amendement n° 80 rectifié . Cet amendement a pour objet d'interdire l'enregistrement des conversations entre un avocat et son client dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. En effet, alors que l'article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l'exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d'écouter et d'enregistrer ces mêmes correspondances. De telles dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l'avocat et aux droits de la défense. Par conséquent, il est proposé, dans le cadre de l'article 100-5 du code de procédure pénale, d'interdire explicitement l'interception et l'enregistrement des échanges

En accordant aux parties le droit d'accéder au dossier avant leur audition ou leur interrogatoire, cet amendement vise à garantir l'effectivité du droit à un procès équitable. Autoriser les parties à accéder au dossier avant leur audition et leur interrogatoire permettrait aux mis en cause de mieux appréhender les accusations portées contre eux et de préparer leurs arguments de défense.

à l'article 114 du code de procédure pénale que le témoin assisté a accès au dossier de la procédure. Je vous le rappelle, l'article 113-3 du même code prévoit déjà un tel accès pour le témoin assisté,

prévoit que les parties ont accès au dossier de la procédure après la réception de la convocation de la première comparution ou audition et donc préalablement à celle-ci. À mon sens, une telle disposition n'est ni souhaitable ni réalisable, l'interrogatoire de première comparution ayant lieu souvent dans le cadre d'une présentation immédiate, à l'issue de la garde à vue. En outre, cet accès, prévu uniquement après l'interrogatoire de première comparution, ne met pas en péril les droits de la défense, la personne pouvant, si elle le souhaite, garder le silence et ainsi attendre d'avoir accès à la procédure pour s'exprimer. Par ailleurs, si un avocat a été désigné et s'il est présent, il aura la possibilité d'avoir accès aux procès-verbaux.